d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. J’informe le Sénat que la liste des candidats proposés par la commission des affaires sociales pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été publiée. Cette liste sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Pour simplifier le calcul des cotisations sociales, en l’établissant sur une assiette unique, et pour améliorer les droits en matière de retraite des exploitants agricoles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Or les dispositions de l’article L. 136 4 du code de la sécurité sociale relatives à l’assiette des exploitants agricoles, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, suscitent de grandes inquiétudes, car elles prévoient une assiette sociale plus large que celle qui est actuellement appliquée. En effet, certains mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits, tels que l’étalement fiscal à court terme de certaines indemnités versées à l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou des subventions d’équipement. Aussi, afin de ne pas pénaliser les exploitants, cet amendement vise à rétablir l’assiette originelle.

de l’assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles, de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus values à court terme réalisées lors de la perception d’indemnités d’assurance à la suite d’un sinistre.

afin de rétablir cette exonération sociale des plus values de cession à court terme exonérées fiscalement, en rétablissant le droit actuellement applicable. L’article 5 ,

à corriger une inégalité de traitement entre nos compatriotes établis hors de France, mise en lumière par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de 2019, qui a sanctionné notre pays.

Cette condition permet d’exclure les investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de la CSG et de la CRDS

J’insiste donc sur un deuxième argument : il n’est pas du tout évident qu’il soit juridiquement possible d’exonérer les Français sans exonérer également les étrangers. Par Par exemple, on peut subordonner l’exonération à l’assujettissement à un régime français obligatoire d’assurance maladie, mais le lien entre cette condition et l’exonération de CSG ou de CRDS n’est pas manifeste. Pour cette raison, il est douteux qu’une telle disposition survive à un recours devant le juge constitutionnel. Pourrons nous vraiment expliquer à nos compatriotes que tel ou tel étranger fortuné, voire très fortuné, est exonéré de CSG et de CRDS sur ses investissements en France ?

auxquelles les Français établis dans ces États tiers sont assujettis, sans pour autant bénéficier des prestations sociales auxquelles ces contributions ouvrent. Ils sont d’ailleurs souvent contraints de s’affilier à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence,

Parallèlement, l’amendement tend à prévoir une légère baisse du taux pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros. Cette mesure répond à un double objectif : renforcer la justice sociale

CSG et de CRDS, soit de 165 euros par mois, ce qui est gigantesque, quand le retraité bénéficie, lui, d’un taux de CSG à 0 % pour une pension au niveau du Smic. L’inégalité va encore plus loin

injuste, ne répondant, selon la Cour des comptes, à aucune logique de politique publique, rapporte 1 000 euros par an à un retraité percevant une pension de 2,5 fois le Smic, comparativement à ce que paie un actif. Je ne vois aucune justification à ce que les retraités, notamment les plus aisés d’entre eux, bénéficient d’une règle dérogatoire au droit commun, alors que notre système social souffre d’un déficit que nous devons absolument résorber. Cet amendement vise donc à aligner le taux de CSG des retraités les plus riches sur celui des actifs, qui sont, eux, tous à la même enseigne. Il s’agit d’un amendement de justice fiscale qui permet de rapporter 1,3 milliard d’euros et ainsi de combler une partie du déficit des branches vieillesse et maladie. Madame la rapporteure générale,

y compris aux revenus de remplacement. Cette mesure visait à améliorer le pouvoir d’achat des actifs en baissant, en échange, les cotisations chômage et maladie et en faisant davantage contribuer les personnes inactives au financement de la protection sociale.

C’est précisément le sens du budget que vous nous présentez. Vous refusez obstinément, de façon idéologique et totalement fermée,

Le scrutin est ouvert.

Je ne vois pas de justification au fait que des gens bénéficiant d’un même niveau de revenu contribuent différemment au financement de la sécurité sociale. Il s’agit du reste d’une entorse à l’exigence de juste répartition fiscale.

fait le choix, dans ce PLFSS, de moduler la revalorisation des pensions en fonction du niveau de vie des retraités.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

48 % entre 2021 et 2023. De fait, sur certains produits, les marges s’établissent entre 30 % et 60 %. Cette boucle prix profit dans le secteur agroalimentaire et les surmarges induites

le Gouvernement a fait une proposition qui vise à instaurer une contribution exceptionnelle temporaire sur les bénéfices des très grandes entreprises. Le dispositif serait ciblé sur les très grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et qui sont redevables de l’impôt

Cet amendement vise donc à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les entreprises pétrolières, afin de financer notre sécurité sociale. En résumé, nous sommes pour l’instauration d’un principe « empoisonneur payeur », afin que la sécurité sociale soit aussi financée par ceux qui nuisent à notre santé. Quel

en difficulté. Mais vous ne voulez pas vous attaquer aux recettes ! Et quand M. Dhersin propose une mesure, somme toute très modérée, qui compense en petite partie une injustice, vous levez les bras au ciel et vous dites

Ils doivent y contribuer de manière progressive, en fonction de leur rémunération. C’est le principe de l’impôt que nous appliquons. L’impôt étant progressif, la participation doit l’être également. Si votre

qui présentent des risques exceptionnels, notamment lorsqu’elles ne respectent pas les règles d’hygiène et de sécurité ou n’observent pas les mesures de prévention édictées par la caisse.

en redéfinissant la répartition des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises donneuses d’ordre. Nous considérons qu’il faut s’inspirer de ce décret pour renforcer la culture de la prévention dans les entreprises

En France, les artistes et les auteurs tirent l’essentiel de leurs revenus du droit d’auteur, qui est défini par le code de la propriété intellectuelle. Une rémunération n’étant pas un salaire à proprement parler, une affiliation des artistes auteurs au régime général a été progressivement mise en place, sur le fondement d’une conversion du montant du droit d’auteur en nombre d’heures au Smic horaire. Mes chers collègues, comme vous le savez, la rémunération de nos artistes auteurs est extrêmement faible. En 2017, 53 % des artistes graphiques et plastiques ont perçu moins de 8 703 euros de revenus artistiques. C’est pourquoi, en 2020, le rapport de Bruno Racine recommandait d’étendre le périmètre des activités accessoires qui leur permettraient d’atteindre plus facilement le seuil d’affiliation Le code de la propriété intellectuelle prévoit explicitement l’existence d’un droit de représentation, qui justifierait de rémunérer les artistes visuels lors des expositions ou les auteurs lors des salons. Cet amendement vise donc à favoriser la rémunération du droit de représentation des artistes auteurs et à aligner son régime social sur celui du droit d’auteur sur la base du barème prévu par le ministère de la culture, même si celui ci n’est toujours pas appliqué.

Mes chers collègues, les réponses du ministère de la culture ne sont pas à la hauteur de la détresse financière des auteurs concernés. En 2017, un dispositif de rachat des trimestres

de diversifier les sources de financement et recommande ainsi de songer à une compensation du manque de cotisations issu du recours à des agents contractuels par l’instauration d’un prélèvement au bénéfice de la CNRACL sur les salaires versés aux agents contractuels.

extrêmement important pour les collectivités locales et les hôpitaux, qui vont voir le taux des cotisations qu’ils versent à la CNRACL augmenter pendant trois ou quatre ans consécutifs,

qui accueillent des établissements sociaux sont en difficulté. Il convient donc de trouver les solutions qui leur permettront d’alléger leurs charges

Il vise à généraliser les possibilités d’exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif. En effet, cette taxe représente une charge significative pour ces établissements, qui emploient un personnel nombreux et spécialisé,

et les organismes d’intérêt général. Les ESSMS, malgré leur mission d’intérêt public, ne bénéficient pas tous de cette exonération

à l’aide sociale, où ils font l’objet d’une gestion administrée et où ils ne fixent pas librement leurs tarifs. De plus, ces deux types de structures sont soumis aux mêmes obligations en matière comptable, à la même gouvernance, aux mêmes conditions de tarification et de contrôle de gestion, aux mêmes règles sociales pour le personnel et à la même réglementation en matière de marché public. Nous demandons donc de rétablir un parallélisme des formes entre Ehpad publics autonomes et Ehpad publics territoriaux.

pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Nous souhaitons ne conserver qu’un taux unique de 4,25 afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de permettre une revalorisation des salaires dans les secteurs sociaux et médico sociaux. J’ajoute que cet amendement a

qu’elle est actuellement conçue, freine le développement de la qualité des prestations et réduit les marges de manœuvre des structures quant à la rémunération de leur encadrement intermédiaire.

salaires, ce qui grève la compétitivité de nos entreprises et empêche les chefs d’entreprise d’augmenter sensiblement les salaires. Nous fonçons dans le mur sans vouloir l’assumer ! La démographie va nous placer dans une situation d’asphyxie financière. Malgré la dernière réforme des retraites, nous nous apercevons que le régime va rester durablement déficitaire et que cela ira de mal en pis. Nous devons donc envisager la piste de l’instauration d’un pilier de retraite par capitalisation.

Actuellement, les retraités américains investissent massivement dans l’économie française par l’intermédiaire de BlackRock, Vanguard ou d’autres sociétés de gestion. Cette situation est absurde, mais elle est bien réelle ! La capitalisation pourrait à la fois permettre de sauver notre système de retraite, d’augmenter durablement le niveau des pensions versées et de faire financer notre économie par de grands fonds de pension qui investiraient dans nos entreprises. Quel

pérennise le dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2025,

il soutient également l’activité économique en zone rurale, car il apporte des bénéfices essentiels aux petites et moyennes exploitations agricoles. Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas aux salariés des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers

amendement vise donc à intégrer les Etarf au dispositif TO DE. Cette mesure paraît pleinement justifiée par la nature saisonnière de leurs activités, qui sont liées aux cycles de la production animale et végétale. Durant ces périodes, les emplois saisonniers représentent près de 70 % de leurs effectifs. Adopter cet amendement reviendrait à renforcer la compétitivité économique de l’agriculture française et à soutenir l’emploi et la pérennité de ces entreprises, qui structurent nos territoires ruraux.

travaux d’amélioration foncière agricole, ainsi qu’aux travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération.

des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois […] sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine

de règles du droit du travail. Cet amendement vise, d’une part, à garantir des conditions de travail à tout le moins décentes des mécanismes de contrôle adaptés et, d’autre part, à assurer le respect du droit au repos hebdomadaire. droit au repos hebdomadaire. Mes chers collègues, je vous rappelle que le Gouvernement a publié, en juillet dernier, un décret permettant aux entreprises agricoles, notamment en Champagne, de déroger à l’obligation d’accorder un jour de repos hebdomadaire. Or ce jour

Il convient de lutter contre ces dérives en réservant le bénéfice de l’exonération TO DE aux employeurs respectant les règles élémentaires du droit du travail.

Nous proposons de soumettre l’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi à l’existence d’un logement digne, à la protection des salariés lors des canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche et à la prise en charge des frais de transport.

initialement pour objectifs d’améliorer la compétitivité des entreprises, de créer de l’emploi et de lutter contre le travail illégal.

réelle évaluation. Le travail saisonnier agricole représente 250 000 à 300 000 salariés chaque année, soit un quart de l’ensemble des contrats saisonniers de notre pays. Le TO DE profite en premier lieu aux filières à haute intensité de main d’œuvre

Les pertes financières sont considérables dans les élevages ovins qui, dans certaines régions, dont la Corse, représentent une activité essentielle pour l’économie locale. En exonérant nos agriculteurs des cotisations sociales, nous leur offrons un répit crucial, une bouffée d’air, alors que les charges s’accumulent que la mortalité des animaux et la baisse de la production compromettent leur avenir. C’est donc une mesure de solidarité, de protection et de soutien envers nos agriculteurs

temporaire, les producteurs agricoles touchés par la crise de la filière de la canne à sucre. Cette exonération s’apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s’appliquerait que pour les rémunérations de l’année 2024.

suscite en effet de nombreux blocages, des manifestations d’agriculteurs, de transporteurs ou de coupeurs de canne, signe de la crise permanente qui frappe cette filière

de la manière que vous voudrez ! Je sais bien qu’il ne faut pas déshabiller la sécurité sociale, mais il ne faut pas non plus tuer les agriculteurs. Je vous en conjure : faites le nécessaire

Les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux sont malheureusement concernées par cet abaissement de l’abattement fiscal de 71 % à 50 %, et l’abattement supplémentaire dont bénéficiaient jusqu’à présent les gîtes ruraux a été supprimé, malgré mes efforts en Du fait de ces modifications, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gîte rural vont se retrouver assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevé.

sociales les revenus qu’ils tirent des activités de location des gîtes ruraux, lorsque les revenus générés bénéficient de l’abattement fiscal en micro BIC prévu à l’article 50 0 du code général des impôts. Quel

complément de ressources et de contrebalancer la variabilité des recettes liées aux productions agricoles. Dès lors, ces revenus sont partie intégrante des produits de l’exploitation

En effet, dans l’ensemble des collectivités d’outre mer, qui sont des territoires éloignés ou insulaires, la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur, lié à l’accompagnement des transitions écologiques et à la garantie d’un revenu décent aux agriculteurs. Or, depuis plusieurs dizaines d’années, en dépit du volontarisme des élus locaux, on assiste à une décroissance significative de la surface agricole utile en Martinique. Le nombre d’exploitations agricoles a en outre connu une baisse drastique, signe d’une concentration des terres et d’un abandon des petites exploitations. Aussi, face à cette crise des vocations,

hectares en moyenne en Martinique –, engendrent trop peu de revenus pour inciter les jeunes générations à s’installer. Pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de notre agriculture, redonner l’envie d’entreprendre, il est donc nécessaire de simplifier le quotidien des jeunes agriculteurs et d’alléger leurs contraintes. Tel est l’objet de cet amendement, inspiré des mesures préconisées

pour les exploitations inférieures à quarante hectares, ce qui concerne 98 % des exploitants agricoles ultramarins. En conséquence, votre amendement doit être rejeté, car il est déjà satisfait.

qui influe fortement sur l’équilibre budgétaire. En effet, il existe de nombreuses exemptions d’assiette sur les cotisations sociales. Ces parts de revenu ne sont pas considérées dans le calcul des montants dus pour les cotisations

protection sociale, que nous défendons : un revenu crée un devoir de cotisation et ouvre un droit à la protection. Ces exemptions multiples et variées ne sont donc pas bienvenues par principe. La diversité des formes d’exemption fait que peu d’évaluations globales ont été menées. Toutefois, le rapport Bozio Wasmer, sur lequel le Gouvernement et la majorité sénatoriale se sont appuyés,

Stéphane Fouassin. L’imbroglio juridique actuel rend illisible le droit social applicable à Mayotte, disséminé à travers des ordonnances, le code de la sécurité sociale applicable à Mayotte, le code de la santé publique et divers autres textes. Ce manque de clarté contribue au ralentissement de la convergence des droits sociaux à Mayotte. Afin d’obtenir une égalité sociale réelle dès 2027, le rapport demandé au travers de cet amendement devra clarifier les écarts de taux existants et les dispositifs applicables, non applicables ou partiellement applicables,

madame Poncet Monge.

: La parole est à M. Éric Gold. Cet amendement est adopté tous les ans au Sénat depuis 2021 avant d’être, chaque fois, sacrifié au cours de la navette parlementaire. Nous espérons que le nouveau gouvernement y sera plus favorable. Notre objectif est toujours de récompenser les collectivités qui s’engagent dans l’action sociale, notamment dans le maintien des personnes à domicile.

Le gouvernement précédent avait à l’époque indiqué vouloir réserver l’exonération aux structures spécialisées. Nous vous proposons donc une exonération pour les EPCI ayant pour objet l’action sociale. Quel est l’avis de la commission ? Avec la même constance, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Merci

place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Voté en 2012 dans le sillage de la crise financière de 2008, le CICE a été créé

Depuis 2019, le CICE a été transformé en exonération pérenne de cotisations sociales pour les entreprises, sans aucune condition.

au traitement des cancers, qui représentent en moyenne 1 500 euros par an. Quel

les organismes mettent eux mêmes en avant. Cette mesure serait sans impact sur les finances publiques dans la mesure où elle sécurise juridiquement une pratique. Le gage n’a donc pas d’autre finalité que de garantir la recevabilité financière de l’amendement et nous appelons le Gouvernement à le lever. Quel

Poly, sur l’article. En 2024, les exonérations et les exemptions de cotisations sociales ont représenté – faut il le rappeler ? – 88 milliards d’euros. Chaque année, le coût des baisses de cotisations sociales augmente de 10 %. Engagée depuis des décennies et maintenue coûte que coûte, comme un mantra, l’augmentation incontrôlée des exonérations de cotisations entraîne un double mouvement d’assèchement des recettes de la sécurité sociale et d’étatisation. Chaque année,

et dénaturent notre modèle de protection sociale. Pourtant, la politique d’exonération de cotisations sociales, justifiée par le « coût du travail », a démontré son inefficacité.

compris entre 1,3 Smic et 1,9 Smic, afin de récupérer 5 milliards d’euros. Pourtant, malgré cet effort apparent, la part des cotisations sociales dans le financement de la sécurité sociale continue de s’effondrer. Néanmoins, nous prenons cet article pour ce qu’il est : un premier pas vers la remise en question des allégements de cotisations sociales. Nous voterons donc pour.

un débat nécessaire, car l’explosion de ces exonérations grève les comptes publics. Actuellement, les exonérations en faveur de l’emploi s’élèvent à près de 91 milliards d’euros. Hors exemptions, elles sont plafonnées

préconisait d’aller plus loin en diminuant les exonérations pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 Smic, ce qui permettrait de dégager 6 milliards d’euros. Nous proposons d’aller encore plus loin plus loin en fixant le point de sortie des exonérations à 2 Smic, ce qui permettrait de dégager 8 milliards d’euros – un montant très précieux pour l’équilibre de nos comptes. Rappelons que la sécurité sociale française repose sur un système simple : le travail crée un devoir de contribution pour la mutualisation des risques et ouvre un droit à la prise en charge solidarisée des aléas de la vie. Les politiques des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont délégitimé ce fonctionnement et fragilisé le principe de solidarité et de mutualisation des risques. Or c’est la base de notre système de sécurité sociale ! Nous voulons trouver l’équilibre, en supprimant les exonérations qui n’ont aucun impact sur l’emploi et sur la compétitivité de nos entreprises. entreprises. Vous l’avez dit, madame la ministre, notre sécurité sociale est un trésor national que nous devons protéger. Pour cela, il nous faut des recettes

D’abord, cette mesure n’améliorera en rien le pouvoir d’achat des salariés. Au contraire, elle entraînera un gel des salaires renforçant ce que vous avez appelé la « smicardisation », c’est à dire une convergence vers le salaire minimum au détriment des revalorisations salariales.

Enfin, il ne faut pas sous estimer l’impact sur le chômage : la hausse des charges pèsera sur la création d’emplois, particulièrement pour les publics les plus vulnérables. Dans un contexte déjà difficile où l’inflation fragilise les entreprises et les ménages, cette réforme pourrait provoquer des fermetures en cascade, aggravant encore la situation économique du pays. Face à ces dangers, il est de notre devoir commun de demander la suppression de cet article. Protégeons nos entreprises, nos emplois et le pouvoir d’achat des Français au lieu d’imposer des réformes idéologiques qui ne servent qu’à remplir temporairement les caisses de l’État au détriment du long terme. L’amendement

ci prévoit de réformer les règles d’allégements généraux de cotisations patronales, ce qui risque d’avoir un impact important sur beaucoup de TPE PME, qui sont dans l’incapacité d’augmenter les salaires au vu des conséquences qu’aurait une telle augmentation sur les prix de vente. Cela enrayerait toute reprise possible de l’activité des entreprises. La réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette du calcul des cotisations sociales serait un autre coup porté aux TPE, car cette prime est aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible aux petites

Il prévoit notamment la baisse de quatre points d’exonération au niveau du Smic. Cette mesure va à l’encontre des politiques de soutien à l’emploi menées depuis 2017, qui ont permis de réduire significativement le coût du travail et de stimuler l’emploi, en particulier pour les petites entreprises. le taux de chômage – vous l’avez rappelé, madame la ministre – n’a jamais été aussi bas depuis quarante ans. Ces politiques d’exonération ont permis de créer 2,5 millions d’emplois depuis 2017. La suppression de certaines de ces exonérations, notamment au niveau du Smic, entraînerait une hausse importante du coût du travail. Elle reviendrait à inverser

Mes chers collègues, pour préserver les acquis en matière de réduction du chômage et de compétitivité, il me semble plus sage de supprimer l’article 6. L’emploi ne peut pas être une variable d’ajustement budgétaire. L’enjeu est clair : maintenir les créations d’emplois, soutenir nos PME et garantir la compétitivité de notre économie. En supprimant le présent article, nous affirmons notre engagement envers une politique économique responsable et sociale. La parole

Ces exonérations sont non pas un privilège, mais un outil vital pour soutenir le tissu économique et social de territoires confrontés à des réalités structurelles bien différentes de celles de l’Hexagone. Notre objectif est clair

Il s’agit d’une proposition équilibrée et responsable. Nous avons également veillé à la soutenabilité financière de la mesure. La perte de recettes pour la sécurité sociale sera intégralement compensée par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Ce choix est pragmatique et juste et ne met pas en péril les comptes sociaux. Mes chers collègues, cet

Merci,